La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

régies par le code de commerce. Nous préférons que le Parlement reste pleinement saisi de ces sujets. Les amendements parlementaires qui visent à étendre un champ d'habilitation à légiférer par ordonnance sont directement contraires au premier alinéa de l'article 38 de la Constitution. Il est donc demandé au Sénat

En l'état, mon groupe ne votera pas cette motion d'irrecevabilité.

Le scrutin est ouvert.

Tout à l'heure, M. le ministre, sans aucune explication, a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 269 rectifié, qui visait à faire figurer une clause imposant le paiement d'un acompte dans la proposition de contrat écrit que l'acheteur doit remettre au vendeur. L'avis du rapporteur fut tout aussi défavorable et le Sénat a décapité l'amendement n° 269

de l'article 152 du règlement Omnibus énonce que « les agriculteurs, incluant les associations d'agriculteurs, et leur premier acheteur peuvent s'entendre sur des clauses de partage de la valeur Comprenez ainsi qu'il ouvre la possibilité aux interprofessions de construire un partage de la valeur ajoutée. Un rôle est également donné aux organisations interprofessionnelles pour établir des clauses standard de partage de la valeur ajoutée. À noter que ce régime a déjà fait ses preuves dans des systèmes de régulation et de gouvernance comme celui du comité interprofessionnel du gruyère et du comté. Le second objectif est de objectif est de rétablir la possibilité, pour les interprofessions, d'intégrer dans les contrats qu'elles proposent des clauses relatives au principe de prix plancher. Néanmoins, nous sommes lucides : un contrat n'a jamais rééquilibré une relation commerciale. Nous restons persuadés que c'est en modifiant les structures de marché que les pouvoirs de négociation peuvent se rééquilibrer. Il est important d'affirmer la nécessité de prix planchers d'achat définis collectivement et prenant directement en compte les coûts de production.

la mission d'« améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché » et, d'autre part, à tirer les leçons de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne relatif au dossier dit du « cartel des endives ». Il tend ainsi à apporter une sécurité juridique indispensable à ces organisations, qui doivent, notamment, pouvoir établir des dispositifs d'échanges d'informations stratégiques- plus particulièrement relatives aux prix et aux volumes des produits mis en marché -, sans craindre d'encourir des sanctions au titre du droit de la concurrence. concurrence. L'argument du droit de la concurrence est trop souvent mis en avant par certains maillons pour ne pas mettre en place des actions à visée économique. Les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir des dispositifs de collecte, d'analyse et de production de données, y compris relatives aux prix et aux volumes, permettant à leurs adhérents de l'amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans les négociations avec leurs acheteurs. Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des indices et l'ancienneté des données utilisées soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir un reflet fidèle

est à M. Michel Vaspart. Sans contester l'utilité et l'importance de la diffusion et de l'élaboration d'indicateurs au sein des organisations interprofessionnelles, il convient d'être vigilant sur le fait que ces indicateurs ne conduisent pas à des actions coordonnées sur les prix qui pourraient placer l'ensemble des acteurs de l'organisation interprofessionnelle dans l'insécurité juridique. Cette problématique a été particulièrement relevée par l'Autorité de la concurrence, dans son avis en date du 3 mai 2018. Cela concerne le contenu des indicateurs- jusqu'où de tels indicateurs peuvent aller -, mais aussi les éventuelles « recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix qui pourraient être effectuées par les organisations interprofessionnelles. Par sécurité juridique, il est préférable de supprimer cette disposition du projet de loi. De plus, le prix doit rester du ressort de la négociation entre les producteurs- organisation de producteurs,

est à M. Claude Bérit-Débat. La rédaction actuelle tend à laisser croire que la répartition de la valeur pourra se décider de manière unilatérale au sein des organisations interprofessionnelles. Dans le cas précis visé par cet alinéa, ce n'est pas l'article 172 du règlement OCM unique qui doit être visé, lequel est relatif à la capacité des agriculteurs et de leurs associations de négocier des clauses de partage de la valeur, mais l'article 157 dudit règlement, qui permet aux organisations interprofessionnelles d'établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l'article 172 . Cette précision a son importance, car ne pas modifier cette rédaction pourrait instaurer un doute, voire une insécurité juridique pour les AOP le texte pourrait être interprété comme permettant aux interprofessions de se substituer aux producteurs eux-mêmes dans la négociation du partage de la valeur. Il importe donc de maintenir la clarté du texte sur ce point et de garantir une bonne répartition des missions incombant aux organisations interprofessionnelles et aux organisations de producteurs, conformément à la réglementation européenne. L'amendement

au sein des filières. Actuellement, la réglementation européenne ne permet pas que ces clauses fassent l'objet d'accords étendus. Toutefois, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire de figer cette impossibilité en l'inscrivant dans la loi. la loi. La réglementation européenne pourrait évoluer sur ce sujet et l'inscription dans notre législation de cette impossibilité formaliserait un cadre trop rigide. La suppression de ces mots n'enlève donc rien à la portée de cet article tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale, car la réglementation européenne reste la même. Ainsi amendé, il permettra en revanche une meilleure adaptation au cadre européen futur. Je précise que nous avons été interpellés par une partie du monde agricole, certains syndicats craignant que cette inscription dans la loi n'envoie un mauvais signal aux interprofessions où l'aval de la filière rechigne déjà à discuter de clauses types de répartition de la valeur. C'est pourquoi nous vous invitons à voter cet amendement.

pas l'obligation et ne sauraient l'avoir, puisque ces organismes privés déterminent eux-mêmes leurs missions. Il est impératif de supprimer la référence au principe de prix planchers dans la loi, puisque l'idée d'une entente des interprofessions sur un prix minimum est contraire au droit de la concurrence européen. Avis défavorable. L'amendement n° 66 pose plusieurs difficultés. Dans le règlement OCM, les missions des interprofessions sont au nombre de quatorze. L'amendement n'en mentionne que deux sur ce total. Il prévoit que les interprofessions peuvent procéder à des échanges d'informations stratégiques. Or cette possibilité est réservée aux seules OP. Avis défavorable. L'amendement n° 293 rectifié rappelle à juste titre que, lors de leur élaboration des indicateurs, les interprofessions doivent effectivement se montrer vigilantes, car ces indicateurs ne doivent pas se transformer en recommandation de prix ou en prix imposé. Tant que les parties sont libres de choisir parmi les indicateurs disponibles pour élaborer leur formule de prix, cela ne pose pas de problème. Il en va de même des recommandations, qui ne sont ici qu'une faculté. Tant que celles-ci ne se transforment pas en une obligation créant une entente sur un prix, il n'y a pas de difficulté avec le droit de la concurrence. Avis défavorable. visent à apporter une clarification rédactionnelle à laquelle je suis favorable.

même si je peux soutenir les propositions consistant à rappeler dans le code rural certaines dispositions du règlement OCM, à savoir la possibilité pour les interprofessions de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ou à élaborer et diffuser des analyses sur les perspectives d'évolution de marché,

le règlement Omnibus n'a pas ajouté les clauses de répartition de la valeur à une liste exhaustive- elles figurent à l'article 164 de l'OCM, qui porte sur les actions pouvant faire l'objet d'un accord interprofessionnel étendu. En conséquence, le règlement Omnibus indique bien que ces clauses ne peuvent faire l'objet d'accords

pour faire monter le pire dans la population agricole de notre pays. Vous m'avez répondu

viticole. Des accords ont été passés entre les différents producteurs, mais, en pratique, les règlements peuvent intervenir à la fin de l'année culturale, par contrat.

à la récolte suivante, en application de la mention « jusqu'à la fin de l'année culturale en cours ». Cette dernière notion couvre l'entier cycle de production jusqu'à la récolte. Comme la facture

monsieur le ministre, l'amendement aurait pour effet de faire passer, pour le secteur vitivinicole, les délais de droit commun de 45 jours à plus d'un an, sans contrôle possible par les autorités compétentes, comme vient de le dire

ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Cet article permet aussi de déroger à ces délais par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture notamment, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs. En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende est prévue pour les personnes physiques, et une amende d'un montant plus élevé pour les personnes morales.

; le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ; toute autre raison objective justifiant la dérogation. La parole

trouvent des vignobles. Il y est fait référence à l'article L. 443-1 du code de commerce, lequel prévoit des dérogations aux délais de paiement contractuels. Ces dérogations peuvent être instaurées par accord interprofessionnel, et sont négociées au sein de chaque interprofession. Pour la filière viticole, le recours à ce régime dérogatoire est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs, ce qui permet de répondre à des contraintes spécifiques de la filière. Dans le cadre de cette procédure d'extension des délais de paiement par accord interprofessionnel, l'autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs. tout le problème réside dans la manière dont l'autorité administrative apprécie le délai fixé par l'accord interprofessionnel. Dès lors, il apparaît important que soit précisé dans la loi ce qu'est un délai de paiement non manifestement abusif. L'amendement tend donc à prévoir que les délais de paiement interprofessionnels soient présumés non abusifs s'ils sont adoptés à l'unanimité des deux familles professionnelles, et que le caractère manifestement abusif des délais de paiement soit apprécié par l'administration au regard d'éléments pertinents, notamment les critères suivants : l'existence éventuelle d'un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux- mauvaise foi et usage déloyal ; les spécificités du secteur et du produit concerné

les réserves présentes dans les caves sont plus importantes, en valeur, que le chiffre d'affaires annuel des négociants ou des

Cet amendement fait écho à la proposition de loi déposée en 2015 par notre collègue député André Chassaigne. déjà fait le constat, à l'époque, de l'inefficacité des négociations ponctuelles intervenant en période de baisse importante des prix d'achat, le plus souvent sur l'initiative du ministre chargé de l'agriculture. Aujourd'hui, le monde agricole partage très largement l'idée selon laquelle il est nécessaire de mettre en place de véritables outils d'intervention sur la fixation des prix d'achat des productions agricoles, avec l'objectif de couvrir les coûts de production constatés et de garantir un revenu décent qui assure la pérennité des exploitations agricoles. C'est pourquoi nous souhaitons, conformément à l'objectif affiché par le Gouvernement, revaloriser le rôle des interprofessions en leur donnant un véritable levier d'action pour agir en matière de prix dans les relations commerciales au sein de chaque filière. Cette forme de régulation interne aux interprofessions permettrait d'amortir les excès auxquels les fluctuations de prix sur les marchés mondiaux et les stratégies de la distribution donnent lieu régulièrement. Le renforcement du cadre de la contractualisation prévu par le présent projet de loi ne peut s'exonérer de la nécessité d'une concertation globale et annuelle sur la situation des prix et des revenus des agriculteurs dans chaque filière. Aussi, nous proposons la mise en place d'une conférence annuelle de filière, regroupant l'ensemble des acteurs des différentes filières : producteurs et organisations agricoles, transformateurs et distributeurs, en élargissant le champ de la représentativité syndicale agricole. Cette conférence ferait état de l'évolution des coûts de production en fonction des bassins de production et des revenus des producteurs de chaque filière agricole, ainsi que des perspectives d'évolution des marchés

la réunion des filières. Nous avons souhaité, après les États généraux de l'alimentation, et après que les filières nous ont adressé

de la Cour de justice de l'Union européenne rendu dans l'affaire du cartel des endiviers. Cet arrêt n'a pas véritablement tranché la question en ce sens, en réservant cette possibilité aux OP

Cette possibilité étant d'application directe, sa traduction dans la loi s'avère donc inutile. L'amendement, en supprimant cet article, vise à lever toute ambiguïté. Ce sujet est quelque peu particulier, puisque l'autorité de la concurrence, au niveau

L'article que propose de supprimer Jean Bizet par le biais de son amendement n'a pas d'utilité particulière. De plus, dans le cas présent, le droit européen est applicable directement. La commission donne donc un avis favorable. Quel est ? Je m'en remets à la sagesse du Sénat. Je suis également d'avis que la portée de l'arrêt « endives », qui est intervenu antérieurement au changement de la réglementation européenne, est plus large que celle de l'article sur lequel nous sommes en train de travailler. rejoins la position du président Jean Bizet : l'article 5 ne reprend pas les conclusions de cet arrêt. Il est vrai que ce sujet n'est pas simple, et nous devons prendre le temps de le traiter dans le cadre des lignes directrices que le Gouvernement établira pour accompagner l'avis de l'Autorité de la concurrence paru en mai dernier. L'article 5 pourrait cependant faire croire, à tort, qu'aucun échange d'informations n'est possible au sein d'une OP qui ne négocie pas les contrats au nom de ses membres. La parole est

parole est à Mme Françoise Gatel. La loi Sapin II a mis fin à tout procédé de cession à titre onéreux de référence laitière, afin d'éviter des dérives liées à la vente de gré à gré entre producteurs. Si on en comprend bien l'esprit, il faut toutefois admettre que, par la même occasion, ce dispositif a mis fin à des systèmes vertueux, qui étaient coconstruits de manière responsable entre des producteurs et des laiteries. Ainsi, depuis la fin des quotas et avant la loi Sapin II, certaines organisations regroupant des producteurs et des laiteries se sont mises en place pour exercer une gestion commune, ce qui a permis de satisfaire les producteurs permis de satisfaire les producteurs tout en évitant la spéculation. La laiterie connaît en effet les volumes à céder et les jeunes à installer, et elle peut, en commun avec les producteurs, définir des règles très transparentes de redistribution et des prix de cession

et vertueux, est interdit, alors qu'il permet de conforter les exploitations, d'optimiser les moyens de production et d'éviter les spéculations. Je ne doute pas, monsieur le

La loi Sapin II, qui n'est pas très ancienne, a prévu la non-commercialisation de ce type de contrat

le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur les dispositions de la loi Sapin II, qui a été votée il y a peu de temps, en 2016. L'article 1 prévoit la répartition des quantités à livrer entre les producteurs qui sont membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et

d'un bassin, localement, les volumes qui ne sont plus produits par les agriculteurs qui partent à la retraite et par les producteurs qui sont en décroissance, en les attribuant à des jeunes sans dépenser un seul centime.

Votre demande peut être complètement satisfaite, et peut même être organisée. Nous sommes en train de travailler sur le fait que les producteurs puissent, à travers leurs OP, prendre leur destin en main.

mais aussi passionné par cette agriculture française qui a le mérite de couvrir la totalité des territoires français, je pense qu'on ne peut pas entrer dans cette logique qui reviendrait à vendre notre âme au diable

peut-être pas aussi rapidement, mais ils le seront indirectement. Ne les incitons pas à dépenser de l'argent ! J'ai eu des débats animés avec différentes OP sur ce sujet. Pour moi, l'affaire doit être classée en ce sens.

assez remarquable, car elle favorise l'installation de jeunes agriculteurs et pratique un prix du lait inégalé par ailleurs. Cela explique qu'il n'y ait jamais de mouvements d'agriculteurs devant cette laiterie, qui est vraiment écoresponsable et socialement responsable.

OP. Je sais qu'il faut lutter contre la spéculation, mais en même temps je regrette que les défauts d'un grand nombre nuisent à la vertu de certains. Le ministre des affaires étrangères a bien rappelé hier au Président de la République qu'il arrivait aussi aux Bretons d'être extrêmement vertueux. C'est un exemple de vertu qui m'amène ici à défendre les producteurs de chez moi.

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 , supprimé en commission par le rapporteur. Cet article visait initialement à s'assurer de la représentation des OP et des AOP les plus représentatives au sein des interprofessions, conformément à une recommandation du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, dans son rapport sur les interprofessions de mars 2017. de mars 2017. Introduit à l'Assemblée nationale, il avait été réécrit par le Gouvernement qui, de ce fait, lui avait apporté son soutien. Il s'inscrivait dans la lignée de la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, qui instaure une présomption de représentativité des organismes professionnels de la production, lorsque des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentant au moins 70 % des voix aux élections des chambres d'agriculture participent à l'organisation interprofessionnelle. Cet article 5 a été supprimé par le rapporteur de la commission des affaires économiques au motif qu'il était satisfait par le droit en vigueur. Nous estimons toutefois qu'il est parfois nécessaire de préciser davantage la loi pour s'assurer que son esprit soit bien préservé. De plus, si le droit en vigueur satisfait notre amendement, mais que, pour autant, son intégration au texte répond à une attente du monde agricole, nous ne voyons pas pourquoi nous nous priverions de son adoption.

Enfin, compte tenu de la combinaison des dispositions de l'article 1, qui inverse la responsabilité de proposer un contrat, et de l'article 5, qui étend les missions des organisations interprofessionnelles à la définition d'indicateurs, nous pensons qu'il est logique d'encourager la présence des OP au sein des interprofessions.

? On est d'accord, le droit n'est pas une science exacte, mais il lui arrive tout de même d'être précis parfois ! Là, on ne doit pas en faire tout à fait la même lecture Il est évident que, sur le fond, les OP et les AOP doivent être présentes au sein des interprofessions, puisqu'elles sont les maillons essentiels de la structuration de l'offre de production agricole. Tout en partageant ce point de vue, pourquoi la commission a-t-elle supprimé cet article ? Pour un motif simple

l'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges se fait par le biais de son comité de pilotage et sous trois mois. La raison première de cet ajout par la commission des affaires économiques était de conforter l'idée qu'il ne s'agissait pas de demander à la puissance publique de fournir des indicateurs, mais bien de laisser la responsabilité aux acteurs économiques et aux filières de les construire. C'est ce que nous souhaitons. Le passage par le comité de pilotage de l'Observatoire ne permet aucunement

qu'il se substitue aux filières. Pour ces raisons, je vous invite à soutenir l'amendement que je viens de vous présenter.

avance qu'il n'y aura pas d'accord interprofessionnel parce que les intérêts seraient contradictoires ! Ce que nous voulons, c'est responsabiliser les acteurs. Or cette déresponsabilisation au profit d'un organisme extérieur me paraît contraire à toute logique à toute logique de discussion profonde dans l'interprofession pour parvenir à des accords. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'amendement du Gouvernement.

présenter l'amendement n° 68. La loi impose aux entreprises de publier leurs comptes. Malheureusement, un certain nombre d'entre elles ne s'y conforment pas et ne procèdent pas à cette publication. Nous pensons qu'une facilitation de la mise en oeuvre de sanctions pourrait les engager à un plus grand respect de cette loi. Nous avons toutes et tous encore en tête le scandale récent de Lactalis et des laits infantiles contaminés à la salmonelle. Je vous rappelle que MM. Nalet et Besnier, respectivement directeur de la communication et PDG de Lactalis, ont indiqué lors de leur audition que la publication des comptes, qui est- j'insiste -une obligation légale, risquerait de les mettre en danger face à leurs concurrents,

ou au ministre de l'agriculture le pouvoir de demander au président du tribunal de commerce l'engagement d'une procédure d'injonction, avec la possibilité pour le juge d'adresser cette injonction dès le premier manquement. La mise en oeuvre de sanctions peut être peut être accélérée afin que les entreprises récalcitrantes se conforment à la loi. L'objectif de ce renforcement de l'application de la loi est, dans le fond, de remédier à un problème important, celui de l'asymétrie de l'information. En effet, le producteur doit pouvoir disposer, lui aussi, d'informations suffisantes sur le distributeur à qui il vend ses produits. C'est pour cela qu'il est essentiel que cette procédure s'applique également aux entreprises de distribution. Notre amendement, s'il ne résout pas totalement l'asymétrie, vise ainsi à remédier au déséquilibre informationnel existant actuellement, et à rééquilibrer le rapport de forces dans les négociations commerciales. La parole

spécifique pour le secteur agricole, en supprimant la condition de répétition du manquement et en prévoyant une alerte par le greffier. Le par l'OFPM est rendu facultatif. L'objectif est bien de restaurer le principe d'une injonction de dépôt des comptes sous astreinte plafonnée à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé en France par la société, spécifiquement dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ce faisant, l'efficacité du dispositif est accrue : d'une part, je le répète, la condition d'un manquement répété, comme préalable l'injonction, est supprimée, et, d'autre part, je le disais, l'amendement tend à prévoir le déclenchement de la procédure en précisant que le greffier alerte le président du tribunal de commerce en cas de non-dépôt des comptes. Je précise par ailleurs que, depuis depuis un an, nous avons réitéré nos demandes auprès des entreprises qui ne déposaient pas leurs comptes. Bien sûr, il ne faut pas hésiter ! Cela a été fait il y a quelque temps avec l'entreprise Lactalis. Il ne suffit pas de le faire une fois, nous les avons invitées à le faire chaque fois

Or certains cas d'entreprises ne publiant pas leurs comptes sont emblématiques et doivent être traités avec réactivité et fermeté. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à donner le pouvoir au ministre de l'économie et au ministre de l'agriculture, à qui est rattaché l'Observatoire des prix et des marges, de demander au président du tribunal de commerce l'engagement d'une procédure d'injonction. Cela permettra d'accélérer la mise en oeuvre de sanctions, afin que les entreprises récalcitrantes se conforment à la loi.

d'une entreprise peut être appliqué à tout moment par le président du tribunal. Le texte actuel du projet de loi précise que cette sanction peut être appliquée en « cas de manquement répété » ; nous n'estimons pas cette précision utile, dès lors qu'il revient au président du tribunal d'apprécier si une sanction est nécessaire ou non. C'est pourquoi notre amendement tend à préciser que le montant de l'astreinte de 2 % du chiffre d'affaires peut s'appliquer en cas de manquement, qu'il soit répété ou non. Une fois encore, si nous souhaitons que cette loi permette de modifier certaines attitudes regrettables, nous devons faire preuve de fermeté.

ne déposant pas ses comptes de le faire, et peut assortir cette injonction de l'astreinte qu'il souhaite après, le cas échéant, en avoir été informé par le greffier. C'est prévu à l'article L. 611-2 du code de commerce. Il peut aussi déjà être saisi par le ministère public pour procéder à la même injonction.

transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits une obligation plus rigoureuse que pour les autres sociétés commerciales soumises à l'obligation de dépôt de comptes. » Je remarque donc une dissonance entre les membres du Gouvernement- cela arrive dans tous les gouvernements, je vous rassure, mais c'est mon rôle de le souligner ce soir. La commission partage l'avis de votre collègue, monsieur le ministre, elle ne voit pas pourquoi, si une entreprise automobile ne dépose pas ses comptes, elle devrait être moins sanctionnée qu'une entreprise agroalimentaire. Partant de ce constat, la commission a proposé une rédaction mesurée ; elle maintient le dispositif général pour toutes les entreprises et prévoit, pour astreindre plus lourdement les entreprises les plus fautives, celles qui commettent des manquements répétés et que nous connaissons bien, puisque les plus visées font partie du secteur agroalimentaire- d'entre elles viennent tout de même de déposer leurs comptes -, que le montant de l'astreinte puisse s'élever à 2 % du chiffre d'affaires, reprenant ainsi exactement l'esprit de la disposition actuelle. Nous proposons donc une progressivité de la sanction, applicable à toutes les entreprises. Je rappelle d'ailleurs que la plupart des entreprises qui ne déposent pas leurs comptes sont des PME ; leur appliquer une astreinte de 2 % dès le premier manquement reviendrait à leur faire porter une contrainte économique majeure, tout cela pour résoudre les cas marginaux de deux ou trois grandes entreprises récalcitrantes

ces choses sont incluses dans l'amendement gouvernemental, que je vous invite à adopter, car il tend à aller plus loin pour améliorer l'effectivité de la disposition et à restaurer le principe d'une injonction de dépôt des comptes sous astreinte plafonnée à 2

Une entreprise, quelle qu'elle soit, doit respecter le droit ! Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut que les comptes

Le scrutin est ouvert.

public que des entreprises ne satisfont pas à une obligation légale élémentaire consistant à déposer leurs comptes, mais on est en train de dire : « C'est comme ça donc nombreux à faire une proposition consistant à dire qu'il faut peut-être augmenter un peu la contrainte, puisque la justice n'est pas en mesure de faire pression seule.

a les moyens techniques et administratifs de répondre à des injonctions, afin de ne pas embêter les plus petites entreprises. Je suis aussi d'accord pour dire que ces dispositions doivent s'appliquer à l'ensemble des entreprises d'une certaine taille et non seulement au secteur agroalimentaire. C'est une question de justice et, je crois, de bon sens.

dispositif d'arbitrage. Cette disposition apporterait une plus grande sécurité juridique à l'article 6, qui renforce l'efficacité de la clause de renégociation. Le terme « équivalent » à l'alinéa 8 introduit une ambiguïté qui est source d'insécurité juridique. Il est préférable de remplacer les termes « un dispositif de médiation équivalent » par les termes « un autre dispositif de médiation », bien clair qu'aucun autre dispositif de médiation ne peut être prévu par le contrat. L'objectif est que, en cas d'échec de la clause de renégociation et avant de saisir un juge,

des produits alimentaires oblige les acteurs à se couvrir. Néanmoins, nous n'apportons pas les mêmes solutions que celles que j'ai entendues en commission. Nous pensons qu'il est important que les acteurs s'organisent et se couvrent par la relation contractuelle. Une clause de révision automatique, même avec des seuils définis par décret, jouerait à la hausse comme à la baisse. Nous ne pouvons pas priver les acteurs de leur liberté contractuelle et de toute marge de manoeuvre efficace pour la révision des prix. Aussi, inscrire une révision automatique du prix uniformiserait le comportement des opérateurs, ce qui présente une perte d'efficience pour les marchés corrélés, au risque de susciter des spirales inflationnistes.

Pour lutter contre la volatilité des prix, les États généraux de l'alimentation, le Gouvernement et l'Assemblée nationale avaient prévu un mécanisme efficace : revoir les modalités de renégociation contractuelle.

des prix. Les professionnels pourraient faire entendre leurs difficultés, parce que le projet de loi renforce la clause de renégociation, avec un délai raccourci d'un mois et une obligation de passer, en cas d'échec, devant le médiateur des relations commerciales agricoles, qui pourra saisir le ministre de l'économie si la clause lui semble déséquilibrée. n'est pas du tout contraire à l'esprit du texte, je vais essayer de vous le démontrer. On l'a vu lors de la crise du beurre, l'année dernière, le refus de la grande distribution de modifier ses prix, prix de la matière première, la crème, avait beaucoup augmenté et connaissait une flambée, a conduit à une pénurie pour les consommateurs. Cette clause entend apporter une réponse à ce problème. J'ai moi-même, voilà quelques années, fait office de médiateur avec le ministre de l'agriculture pour un certain nombre de produits dont la grande distribution refusait d'augmenter le prix, alors qu'il y avait une forte augmentation du cours de la matière première. On connaît tout de même leur fonctionnement ... La commission a prévu un mécanisme simple et circonscrit strictement aux produits dont le prix est

précision -, la clause de révision s'appliquera bien sûr à la baisse pour coller le plus possible aux prix qui fluctuent sur des marchés volatils. J'ajoute qu'il s'agit bien d'une révision de prix et non d'une renégociation,

Définir les conditions de départ, améliorer l'information et la transparence dans la redistribution des gains et prévoir des modalités de contrôle et des sanctions pour rendre les dispositions plus efficaces

Pourtant, en l'état, la rénovation du cadre contractuel pour le secteur agricole, qui est la finalité principale de ce projet de loi, ne s'applique pas à nos 2 600 coopératives

La suppression de ce dispositif prive aussi les associés-coopérateurs d'une information plus transparente et de conditions de départ facilitées. Nous prenons nos responsabilités. Oui, effectivement, durant les États généraux de

de l'ensemble des parties prenantes, avant de proposer des mesures concrètes, qui seront évaluées au travers d'une étude d'impact. Mes chers collègues, légiférer par ordonnances- j'entends bien ici un certain nombre de récriminations, et je les comprends parfois parfois -n'est pas un déni de démocratie. Au contraire, nous débattons ce soir des termes de ces ordonnances, et nous devrons les ratifier le moment venu. Compte tenu de l'intérêt que nous portons aux coopératives, je pense que nous devrions suivre la démarche du Gouvernement. est tout à fait hostile à l'idée de voter une loi d'habilitation à légiférer par ordonnances pour remettre en chantier l'organisation des coopératives agricoles. Pourquoi ?

Monsieur le ministre, vous avez parlé la plus claire possible, sur les prix de cession des produits agricoles. Il est donc légitime à un moment donné que l'associé-coopérateur dispose d'éléments transparents sur la formation des prix, comme le producteur qui livre dans un cadre non coopératif. L'ordonnance vise à envisager des dispositions pour améliorer l'accès à l'information des associés-coopérateurs sur les relations économiques qu'ils ont nouées avec la coopérative dont ils sont membres. Le système coopératif repose sur la détermination du prix en fin de campagne, en tenant compte de la restriction pour une coopérative à aller s'approvisionner au-delà de ses seuls membres. Il s'agit ici d'examiner la manière dont nous pouvons

des résultats, et le tout, bien évidemment, sans porter atteinte au statut de la coopération auquel, je le rappelle, nous sommes très attachés.

n'arrive pas à comprendre que l'on puisse aujourd'hui mettre en accusation la transparence des coopératives. Premièrement, nul n'est obligé d'adhérer

dit ! Elles permettent au milieu agricole de continuer à se développer, y compris au travers de politiques très innovantes. Pourquoi voulez-vous y toucher ? Pourquoi parlez-vous de transparence ? Comme cela vient d'être dit, il n'y a pas de problème de dépôt des comptes :

de vote. Je voudrais éclairer le débat sous un jour un petit peu différent. Le premier à utiliser la transparence des coopératives, c'est le négoce, qui s'aligne sur les prix de la coopération

c'est l'assemblée générale d'une coopérative qui clôture les comptes et donne le prix définitif payé aux coopérateurs. Ce n'est pas un acompte au mois le mois ; c'est l'assemblée générale qui, elle seule, est capable d'établir le compte final et le prix final payé aux producteurs-

Des femmes et des hommes décident d'adhérer ou non à une coopérative. Ils décident en connaissance de cause, en fonction des statuts ; il y a des règles.

Madame la présidente de la commission, vous avez fait une

d'origine, en assurant le respect du principe de transparence envers les associés coopérateurs. Si le conseil d'administration ou les instances dirigeantes de la coopérative souhaitent diversifier le portefeuille d'activités de la coopérative, en créant une ou plusieurs filiales, ou en prenant des participations dans une société extérieure, ils doivent en référer à l'ensemble des associés. Ces choix stratégiques doivent être connus et leurs conséquences comprises par l'ensemble des associés coopérateurs. La transparence des coopératives est un enjeu majeur de démocratie interne pour ces structures.

et des méthodes plus durables et visent l'amélioration des approches et des services écosystémiques. Le Gouvernement souhaitait la suppression de l'article 8 AA, mais n'a pas été suivi. J'ai déjà indiqué les raisons

plus encore, de la répartition de la valeur. On devrait aussi évoquer la question de la reconnaissance de la valeur intrinsèque des services rendus par l'agriculture à la société dans son ensemble.

pour expérimenter ce que pourrait être le contenu concret de cette prestation. Je voudrais vous donner un exemple pris dans mon département. Une entreprise,

Cette entreprise vient de mettre au point une prestation pour services environnementaux. Elle paie à ses « apporteurs », à ses agriculteurs producteurs de maïs, qui sont au nombre de deux cents, une prestation de 90 euros par hectare,

à ses services de recherche spécialisés, mette en oeuvre cette prestation pour services environnementaux. Les zones de montagne, comme les zones qui sortent de la carte des zones défavorisées,

supprimé par le rapporteur en commission, et qui vise à reconnaître les conventions tripartites dans la loi. Le développement de ce type de convention ou des contrats dits « tripartites » rencontre actuellement un réel succès. engageant les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, ces contrats permettent aux différents acteurs de s'engager sur des volumes et des prix à partir d'un cahier des charges commun. Ils permettent ainsi de s'assurer de la qualité du produit, ce cahier des charges, tout en sécurisant les acteurs par un engagement pluriannuel sur les volumes. En d'autres termes, ce type de contrat permet également d'assurer une meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les différents acteurs, ce qui est- nous semble-t-il -l'objectif du présent projet de loi. Par notre amendement, nous souhaitons apporter une reconnaissance législative à ce type de démarche vertueuse. En commission, cet article a été supprimé au motif qu'il ne fallait pas imposer un cadre trop rigide.

fragiliser ces contrats, mais, aujourd'hui, il me semble que les réserves qui existaient au regard du droit de la concurrence ont été levées. Au mois de mai dernier, l'Autorité de la concurrence a en effet confirmé la légalité de ces contrats- contrats- dans des conditions certes précises, mais qu'il suffit d'examiner. Dans plusieurs pays européens, tels que l'Allemagne, à laquelle il est souvent fait référence, ou l'Italie, les accords entre producteurs, transformateurs et acheteurs contribuent fortement à une meilleure structuration des filières. Dans notre pays, ces conventions rencontrent un engouement depuis quelques années, en particulier dans le secteur du lait. Chacun a pu l'observer. De grands distributeurs ont mis en place ce type de contrat, engage tous les partenaires dans des démarches de qualité et de plus juste rémunération. C'est ce que nous voulons, et c'est l'essence même de ce texte. Aussi, nous pensons que les conventions tripartites sont vraiment un outil profitable

ne posaient, sous certaines conditions, aucune difficulté au regard du droit de la concurrence, cela n'était plus le cas dès lors que de tels contrats venaient protéger spécifiquement certains territoires, ce qui serait évidemment le cas ici. Ce n'est pas

Monsieur le ministre, j'entends toute l'attention bienveillante que le gouvernement auquel vous appartenez porte à l'économie ultramarine. J'en accepte le principe, mais l'amendement de ma collègue répond à une philosophie que je défends personnellement depuis des années : la notion de différenciation territoriale. Le droit n'est pas figé. Notre rôle, c'est de le faire évoluer. Je ne comprends pas en quoi l'amendement de Mme Jasmin pourrait porter un quelconque préjudice si le choix que ma collègue défend correspond à des réalités ultramarines, qui sont partagées

L'article 24 de la loi de finances pour 2018 entraîne de manière incidente une concentration des exploitations agricoles en doublant les seuils prévus à l'article 75 du code général des impôts, qui autorise un exploitant agricole à passer des recettes commerciales en bénéfices agricoles. Ces revenus autres qu'agricoles compensent la fluctuation des revenus des productions agricoles, liée à la volatilité des prix, aux aléas sanitaires et climatiques. Si ces revenus sont indispensables dans beaucoup d'exploitations agricoles et en ont sauvé de nombreuses, à la suite de la chute des rendements des céréales, du prix du lait ou de la viande, cette disposition du code général des impôts entre en contradiction avec les conclusions de l'article 14 des États généraux de l'alimentation, qui préconisent la mutualisation des investissements sous toutes leurs formes pour accélérer la diffusion des innovations de l'agriculture

d'occupation des territoires et peut entraîner un recul de l'emploi, ce qui est évidemment contraire à tous les efforts conduits ces dernières années en matière de lutte contre le chômage. C'est pourquoi le présent amendement vise à revenir à la rédaction antérieure de l'article 75 du code général des impôts. J'ajoute que ce dispositif

aux animaux de compagnie. La rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat soulève plusieurs difficultés : elle ne vise que les produits relevant de la convention unique, ce qui laisse de côté les marques de distributeurs- les MDD -et les produits donnant lieu à une convention particulière elle a recours à des notions de « valeur » et de « volume », qui, dans une rédaction juridique, ne sont pas suffisamment précises ; elle prévoit des modalités d'entrée en vigueur inadaptées- il suffirait aux opérateurs de la grande distribution qui souhaiteraient se soustraire du dispositif d'encadrement des promotions de conclure les conventions avant le 1 mars 2019. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif n'est donc ni opérationnel ni contrôlable et entraînerait une forte insécurité juridique. Le Gouvernement considère que le traitement de manière exhaustive, efficace et concertée des spécificités techniques de l'encadrement des promotions, outre l'examen du texte par le Conseil d'État, implique le recours à une ordonnance, ce qui constitue un

est à M. Claude Bérit-Débat. Si la proposition d'inscrire dans la loi- plutôt que par ordonnance -l'encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir, elle doit être complète et ne pas omettre certains produits. de l'alimentation avaient préconisé un encadrement des promotions de tous les produits alimentaires, y compris les marques de distributeurs, la rédaction actuelle n'encadre que les produits à marque. Or c'est là un élément central des stratégies commerciales déployées par les grandes et moyennes surfaces, pour qui ces produits sont souvent un outil promotionnel primordial. primordial. L'encadrement des nouveaux instruments promotionnels est primordial, mais il ne sera suffisant que si ces produits sont pris en compte et si le dispositif proposé ne peut être contourné. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion- un quart du total. à mon sens, pleinement satisfaisant du point de vue des distributeurs. Cet amendement tend donc à revoir ces deux éléments, en renvoyant la rédaction précise de l'encadrement des promotions à un décret en Conseil d'État.

Or le prix bas n'est pas un juste prix. Le débat public sur le pouvoir d'achat des ménages se focalise sur la recherche des prix bas, y compris pour la consommation alimentaire, en lieu et place d'une véritable politique d'augmentation du pouvoir d'achat. Cela se fait au détriment du revenu paysan, de la qualité, de la traçabilité, de la sécurité sanitaire de notre agriculture. L'encadrement le plus strict des offres promotionnelles est donc nécessaire.

Si, véritablement, la volonté du Gouvernement est d'encadrer aussi les offres promotionnelles décidées et accordées par les distributeurs, cela doit apparaître. L'amendement n° 286 rectifié, présenté

amendements qui viennent d'être défendus, mais votre commission des affaires économiques, mes chers collègues, a décidé de transformer en dispositions d'application directe l'article 9, qui prévoyait le recours à des ordonnances pour relever le seuil de revente à perte et limiter les avantages promotionnels. Afin de donner la portée la plus large possible au dispositif d'encadrement des promotions et de lever toute ambiguïté sur son champ d'application, cet amendement tend à apporter s'applique expressément à tous les avantages promotionnels, qu'il s'agisse de nouveaux instruments promotionnels- les NIP -ou non, qu'ils présentent un caractère instantané ou différé- afin de prendre en considération les fameuses pratiques de « cagnottage » -ou qu'ils soient financés par le fournisseur ou le distributeur. D'autre part, il s'applique tant aux produits alimentaires sous marques de producteurs qu'aux fameuses MDD.

parole est à M. Henri Cabanel. Cet amendement reprend une proposition émise par les députés socialistes ultramarins. Il vise à rendre applicable le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l'article 9 la proposition à l'Assemblée nationale, Mme Ericka Bareigts, ces départements sont confrontés à un phénomène particulier. Sur ces marchés ultramarins, les prix de distribution de certains produits alimentaires dits de « dégagement » sont très inférieurs aux prix pratiqués dans l'Hexagone. Ces produits de moindre qualité, vendus à des prix défiant toute concurrence, inondent le marché et sont achetés par des personnes n'ayant pas les moyens de payer des produits plus onéreux. Cette pratique nuit évidemment aux producteurs locaux, qui voient le marché brutalement submergé par des produits identiques aux leurs, mais à des prix bien inférieurs. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de préciser dans la loi que le relèvement du seuil de revente à perte sera applicable dans les départements ultramarins.

pu être mis en oeuvre et leurs critères d'application ne semblent pas adaptés. Du fait de cette situation et de la persistance des préoccupations, le Gouvernement a demandé à l'Autorité de la concurrence une expertise approfondie des marchés de dégagement.

une telle mesure serait totalement inutile, toutes les informations disponibles à ce jour tendant à montrer que les produits de dégagement ne sont pas revendus à perte. D'autre part, elle risquerait d'être très coûteuse pour les consommateurs ultramarins. L'effet prix du relèvement du SRP

Par ailleurs, l'effort de meilleure répartition de la valeur au plan national doit pouvoir bénéficier aussi aux acteurs locaux des outre-mer, et ce même si le relèvement du SRP ne s'y applique pas. La production agricole locale ultramarine ne représente qu'une très faible part de la totalité des achats de la grande distribution. Il faudra y remédier. Il y a des débouchés commerciaux à aller chercher, mais il nous faut également structurer l'offre et massifier la production. La grande distribution n'a donc pas besoin

terme, monsieur le rapporteur En vertu de l'article L. 442-2 du code de commerce, qui n'est pas remis en cause par l'article 9 du projet de loi, la revente à perte consiste en la revente à un prix inférieur au prix d'achat effectif d'un produit. La réforme

sont les seuls agents économiques susceptibles de vendre leur production à perte. Avec cet amendement d'appel, nous souhaitons mettre en lumière les limites du projet de loi, qui ne permet pas l'interdiction d'un achat à perte. Or trop souvent, pour survivre, l'agriculteur est conduit à vendre à perte, au risque de voir la pérennité même de son exploitation remise en cause. La logique actuelle présuppose que le travail de l'homme peut être sous-payé, mais que les marges des opérateurs de la grande distribution ne doivent pas pâtir de la guerre des prix. En plus de s'apparenter à du dumping social, la vente à perte a des effets néfastes sur le secteur agricole, dont des pans entiers se trouvent menacés, et sur l'économie du pays. du pays. Interdire l'achat à perte, ce n'est pas porter atteinte à la loi du marché ; c'est la rétablir ! Dans la mesure où celle-ci découle du climat de concurrence déloyale entre grands distributeurs, elle entrave effectivement la compétition du marché, plus qu'elle ne la stimule. Sans mesures répressives mettant fin de manière unilatérale aux pressions exercées par les distributeurs sur leurs fournisseurs, la grande distribution continuera de faire la loi et de s'accaparer les marges des producteurs. Les mesures mises en place pour limiter la guerre des prix entre distributeurs, notamment le relèvement du seuil de revente à perte et la mise en place d'indicateurs de prix, ne s'accompagneront pas de revenus plus justes pour les producteurs, si elles ne font pas partie d'un mécanisme global, garantissant que la hausse des prix de distributeurs à consommateurs soit répercutée sur une hausse des prix de producteurs à distributeurs. Par la mise en place de sanctions pour les opérateurs ayant acheté un produit agricole en l'état, à un prix inférieur à son prix de revient effectif, cet amendement vise à assurer une meilleure répartition de la valeur. L'amendement

Dans ce dernier cas, il s'agit plus exactement de « revente » à perte, interdite pour les commerçants et dont le présent projet de loi va relever le seuil de 10 %. En revanche, la vente à perte par un fabricant peut être légale si elle ne tombe pas sous la qualification de la pratique de prix abusivement bas. L'article L. 410-2 du code de commerce précise que, sauf exceptions prévues par la loi, les prix sont « librement déterminés par le jeu de la concurrence ». En cas de situation particulière, « un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix L'amendement vise à tester l'introduction d'un seuil de vente à perte déterminé à partir du coût de production. L'existence d'un tel seuil permettrait de protéger davantage les producteurs de la pression excessive de certains distributeurs. Cette expérimentation donnerait des éléments objectifs d'appréciation des freins ou apports éventuels de l'existence d'un seuil de vente à perte et permettrait de dépasser le débat opposant libre marché et prix administrés. L'ambition portée lors des États généraux de l'alimentation doit se concrétiser par des mesures fortes dans ce projet de loi. Cette expérimentation doit en faire partie. Quel

le seuil de revente à perte. Elle reviendrait sur le principe de la liberté des prix, qui prévaut depuis 1986 et est imposé par le droit de l'Union européenne, pour aller vers un régime rigide de fixation de prix.

présenter l'amendement n° 74. Cet amendement a pour objet d'interdire l'utilisation du terme « gratuit » ou de ses dérivés et synonymes comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale liée à la vente d'un produit alimentaire. En effet, un produit « gratuit » est un produit débarrassé de son prix, mais pas de son coût L'emploi d'un tel terme nie la valeur intrinsèque du produit, des matières premières, éventuellement des animaux impliqués dans le processus de production. Mais employer ce terme, c'est surtout voire dégrader le travail des hommes et des femmes ayant permis la création du produit, ainsi que celui des générations précédentes, qui ont construit notre patrimoine agricole. Cet amendement s'inscrit dans la mécanique globale du présent projet de loi, puisqu'il vise à interdire des pratiques se trouvant aux antipodes de son objectif principal,

Sans reconnaissance sociale du travail des producteurs, aucune reconnaissance économique n'est possible ! Cet amendement vise donc à compléter la mise en place d'indicateurs de prix, afin de garantir un partage équitable de la valeur.

revêt donc un caractère trompeur en termes d'information du consommateur. Si l'utilisation du mot « gratuit » peut déjà être sanctionnée lorsqu'elle relève de pratiques commerciales trompeuses,

présenter l'amendement n° 238 rectifié. Cet amendement vise à rétablir un article introduit à l'Assemblée nationale, qui interdit l'utilisation du terme « gratuité », dans le cadre d'une relation commerciale, par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire. En effet, l'utilisation de ce terme ne permet pas de reconnaître à sa juste valeur le travail fourni par les agriculteurs. cette interdiction permettra aux consommateurs d'avoir mieux conscience de la valeur intrinsèque du produit agricole et de son coût de production. Le mot « gratuité » ne correspond pas à la réalité du processus de production d'un produit, il s'agit, pour moi, d'un mauvais signal envoyé aux producteurs.

élevées ou travaillées par un producteur, il ne peut être considéré comme gratuit. Un aliment a une valeur intrinsèque et un coût de production. Nous sommes peut-être dans le domaine du symbole, mais les mots ont leur importance, à l'heure où nombre nombre d'agriculteurs ne se sentent pas considérés pour leur travail. Il convient certes d'agir concrètement pour leur redonner du revenu, mais aussi de changer nos représentations collectives sur le vrai prix,

gratuitement. Si nous voulons redonner de la valeur à nos produits, notamment pour nos producteurs, nous devons également agir sur les consciences des consommateurs.

faire croire aux gens que des produits sont gratuits à l'achat, c'est leur faire croire qu'ils ne coûtent rien à la production ni aux producteurs et qu'ils n'ont donc pas de valeur intrinsèque. Le débat a eu lieu en commission, et, comme l'a dit notre collègue Joël Labbé, le rapporteur a fait le choix de supprimer cet article au motif qu'il risquait d'être aisément contourné par le recours à des formules moins implicites, mais véhiculant la même idée. Nous pouvons en effet considérer que des stratagèmes permettront de passer outre ce type d'interdiction, mais, pour autant, ne rien faire ne permettrait pas non plus de limiter ce type de promotions dommageables pour les producteurs. Il a été également invoqué, à juste titre, que l'article L. 121-2 du code de la consommation peut déjà sanctionner la mise en avant d'une gratuité dès lors qu'elle induirait le consommateur en erreur au titre des pratiques commerciales trompeuses. Or ce n'est pas l'objet de cet amendement

toutes ont formulé une demande très forte d'encadrement des promotions, ce que prévoit le projet de loi. Ainsi, lorsque le terme « gratuit » ou un terme approchant est utilisé de manière abusive ou trompeuse pour le consommateur, ces pratiques sont susceptibles de faire l'objet de poursuites,

les services vérifient précisément si le consommateur est susceptible d'être abusé par l'information qui lui est donnée ou l'outil marketing qui est utilisé. Il vaut donc mieux travailler sur un bon encadrement des promotions, sur un relèvement du seuil de vente à perte

qui ne sont pas sans incidence sur la préservation de l'image et la notoriété de produits à haute valeur ajoutée. L'article 9 du projet de loi prévoit une disposition habilitant le Gouvernement à renforcer par voie d'ordonnance les dispositions encadrant les promotions afin de lutter contre certaines pratiques excessives. Toutefois, sans assurance sur le contenu de l'ordonnance en matière de pratiques tarifaires pour assurer une régulation économique efficiente et une protection des consommateurs efficace, le présent amendement vise à sanctionner les pratiques réputées abusives en engageant la responsabilité des opérateurs.